Je rappelle que 40 % du suivi des grossesses est actuellement assuré par une sage-femme et que ce chiffre est en constante augmentation du fait de la démographie décroissante des gynécologues obstétriciens. Les sages-femmes assurent déjà le suivi des grossesses physiologiques, le suivi gynécologique de prévention et les interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses et instrumentales. Pourtant, lorsqu'une patiente présente une fausse couche, la sage-femme n'est pas habilitée à lui administrer les médicaments adéquats, car les textes n'ont pas évolué en même temps que ceux qui concernent l'IVG. Une sage-femme peut donc administrer les médicaments appropriés lorsque la patiente décide elle-même d'interrompre sa grossesse, dans le cas d'une IVG médicamenteuse, mais il n'est pas possible de le faire lorsqu'il s'agit d'une fausse couche, alors même que les médicaments sont identiques et à la disposition de la sage-femme. Cette situation accroît l'angoisse des patientes, redirigées vers les urgences, et crée un surcoût pour la sécurité sociale. S'il était adopté, cet amendement permettrait une meilleure prise en charge des personnes concernées

porte ses fruits puisque de nombreuses compétences supplémentaires leur sont dévolues, ce qui est une reconnaissance. Néanmoins, nous regrettons, comme je l'ai indiqué en discussion générale, que l'addition de nouvelles compétences ne fasse pas l'objet, en parallèle, d'une revalorisation de leur rémunération. Nous espérons donc que des négociations salariales seront prochainement menées avec le ministère de la santé et que le en maïeutique sera relevé pour faire face aux besoins actuels et futurs. En attendant, cet amendement, qui est proche de celui que vient de présenter ma collègue centriste, reprend une proposition de l'Union nationale et syndicale des sages-femmes (UNSSF) afin que l'interruption spontanée de grossesse soit traitée par la profession. Les sages-femmes ne doivent pas être limitées à un rôle de prescription de l'accompagnement psychologique : elles doivent véritablement prendre en charge dans

que ce taux est en augmentation : assurant le suivi des grossesses physiologiques, le suivi gynécologique de prévention et les IVG alors que la démographie gynéco-médicale ne fait que fondre à vue d'oeil,

une telle extension doit, selon nous, faire l'objet d'une réflexion plus approfondie. Si les sages-femmes sont, depuis 2016, compétentes pour prendre en charge les IVG médicamenteuses, comme vous le souligniez, elles ne sont toutefois pas autorisées à pratiquer les interruptions de grossesse pour motif médical, l'article L. 2213-3 du code de la santé publique. De plus, elles ne sont autorisées à pratiquer des IVG instrumentales qu'à titre expérimental, après avoir suivi une formation théorique obligatoire ainsi qu'une formation pratique consistant en l'observation de trente actes d'IVG instrumentale et en la réalisation de trente autres. Par ailleurs, les interruptions spontanées de grossesse trouvant souvent leur origine dans une anomalie embryonnaire ou dans des problèmes de santé de la mère, un diagnostic médical peut s'avérer nécessaire, ce que ne peut assurer une sage-femme. Dans ces conditions, il semble précipité de légiférer sur ce point en ouvrant aux sages-femmes une compétence inconditionnelle à prendre en charge les interruptions spontanées de grossesse. Cette question mérite d'être approfondie à l'occasion d'un prochain texte afin d'établir les conditions dans lesquelles les sages-femmes pourront être davantage impliquées dans la prise en charge des patientes.

Je précise que leur statut a été revalorisé à l'occasion du Ségur de la santé puisqu'elles ont vu leurs revenus augmenter de 500 euros mensuels. Néanmoins, comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, ces amendements dépassent le champ des compétences

de la mère. Je reprends le code de la santé publique : l'article L. 4151-3 indique très clairement qu'« en cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, [ ...] la sage-femme doit faire appel à un médecin ». Il faut rappeler

bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché uniquement pour les IVG médicamenteuses. Il n'est possible de le prescrire

approfondi, c'est-à-dire qu'il faut consulter l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités sanitaires, et envisager un complément de formation pour les sages-femmes. Au vu de tous ces éléments, l'avis du Gouvernement est défavorable sur ces amendements.

la grossesse physiologique ou la fausse couche nécessite un diagnostic médical. Cette capacité d'orientation fait partie

ne sont même pas diagnostiquées, parce que très précoces, et sont considérées comme un simple retard de règles par la patiente, qui n'a même pas fait son propre diagnostic de grossesse. Si la fausse couche

Le scrutin est clos.

Ces derniers sont effectivement susceptibles de contribuer à l'accompagnement des patientes connaissant une fausse couche, car certaines femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse se présentent aux urgences sans être systématiquement orientées par la suite dans un service de maternité et gynécologie. Elles

de la commission ? Dans la mesure où les IPA exerçant au sein des services d'urgences sont moins directement impliqués dans la prise en charge des interruptions spontanées de grossesse,

Un arrêté du 25 octobre 2021 mentionne bien la « gynéco-obstétrique » comme motif de recours, mais uniquement pour la c'est-à-dire pour des saignements de l'utérus non causés par une tumeur, une infection ou une grossesse, ce qui ne couvre pas le champ des interruptions spontanées de grossesse.

de suivi psychologique et médical des patientes et de leur partenaire éventuel. Cet amendement tend à préciser l'objectif d'amélioration du suivi médical dans ce parcours en indiquant que la patiente doit obligatoirement se voir proposer un nouvel examen dans les quatre semaines qui suivent l'interruption spontanée de grossesse. Actuellement, à l'issue d'une fausse couche, et dans les cas nécessitant une prise en charge médicale, les femmes sont systématiquement revues en consultation selon les recommandations de bonnes pratiques du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Le nombre de rendez-vous est adapté à chaque situation, à l'appréciation du corps médical. Cet amendement vise à asseoir cette recommandation dans la loi. Quel

C'est pourquoi cet amendement nous paraît contraindre inutilement les praticiens, qui sont les mieux placés pour juger si un nouvel examen est nécessaire. La commission a d'ailleurs, pour ces raisons, supprimé l'article 1 , qui comportait à l'origine cette obligation. En conséquence, nous demandons le retrait de l'amendement

tue -et tant les couples que les femmes seules y sont souvent peu préparés. Il est donc nécessaire d'améliorer l'information sur ce sujet, de l'actualiser annuellement et de la transmettre à un maximum de personnes. Plus les femmes et les couples seront informés des pertes de grossesse précoces, moins ces pertes seront vécues de façon isolée et solitaire ; l'objectif de l'information est de lever progressivement le non-dit et

de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), où l'on peut trouver des précisions sur la définition, les causes et les symptômes des fausses couches, mais aussi un certain nombre de conseils, en particulier celui de s'adresser à un médecin. Je suis donc défavorable à cet amendement. Je précise néanmoins que tout ce qui pourra être fait pour améliorer l'information

Cet amendement vise à renforcer l'information relative aux fausses couches. Environ une grossesse sur quatre trouve une telle fin ; une femme sur dix fait une fausse couche dans sa vie. Au vu de ces statistiques très élevées et du nombre important de femmes concernées, pourquoi attendre que la fausse couche survienne pour en parler ? La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à favoriser l'accompagnement des couples confrontés à une fausse couche ; l'ensemble de ses articles

mon initiative, les objectifs d'information assignés aux « parcours interruption spontanée de grossesse » ont ainsi été étendus et précisés en commission. Toutefois, instaurer une obligation générale et absolue de mentionner les risques liés à la grossesse et, notamment, l'interruption spontanée de grossesse dans le cadre de l'entretien prénatal n'est pas apparu adéquat à la commission, eu égard à la diversité des situations et des vécus des femmes enceintes. La commission a ainsi estimé qu'il revenait au professionnel de santé de déterminer librement s'il était opportun de mentionner ces risques dans le cadre de l'entretien prénatal, en fonction de sa patiente. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. Quel est

sont peu appliquées- dans seulement 15 % des établissements scolaires. C'est pourquoi nous avons fait figurer cette mesure dans le plan « Toutes et tous égaux » que j'ai présenté en Conseil des ministres le 8 mars

Le souhait du Gouvernement est évidemment que la suppression du délai de carence puisse bénéficier à toutes les femmes, sans distinction. Je me réjouis de l'adoption en commission d'un amendement tendant à étendre le bénéfice de cette mesure aux travailleuses indépendantes,

tout, un véritable tabou en France. Pour les futurs parents, cette épreuve est souvent un drame silencieux dont les douleurs sont vécues dans l'ombre. Nous l'avons dit, un mois après l'interruption spontanée de leur grossesse, 24 % des femmes souffrent d'une anxiété modérée à sévère ; 11 % d'entre S'il ne faut ni généraliser les douleurs ni dramatiser les expériences, il n'en demeure pas moins nécessaire d'informer et d'accompagner les couples, et en particulier les femmes ; je pense que cela fait l'unanimité sur nos travées. L'accompagnement psychologique est un premier pas ; nous proposons de lui associer l'ouverture d'un congé spécifique de trois jours pour la survenue d'une fausse couche, à destination de la mère ou des parents concernés. Ce congé serait un moyen de

Y ajouter un congé en cas de survenue d'une fausse couche nous paraît donc possible, utile et nécessaire. Dans la mesure où ce congé serait ouvert autant pour la femme que pour son ou sa partenaire, il ne créerait pas de risque de discrimination pour les femmes, mais permettrait d'offrir aux personnes affectées un peu de remettre, physiquement sinon mentalement. Enfin, ce congé favoriserait l'avancée vers une plus grande égalité au sein du couple et une déconstruction des rôles et des tâches, en permettant au conjoint, quel que soit son genre ou son statut, de s'impliquer tout au long des événements liés à la grossesse et de se sentir directement concerné

Pourtant, aujourd'hui, en France, une femme qui a subi une fausse couche doit prétendre être malade si elle veut se reposer, car elle n'a qu'une option : l'arrêt maladie. Cette fausse assimilation de la

Depuis peu, un tel congé figure aussi dans une convention collective en France, la convention Syntec. Nous proposons donc de modifier la loi pour permettre à toutes les femmes salariées de demander ce congé spécial après une fausse couche.

à son juste titre : ce n'est pas une maladie au sens propre du terme, sauf cas exceptionnel, mais une perte. Certes, des femmes préféreront bénéficier d'un congé maladie par souhait de ne pas révéler leur grossesse cela peut évidemment se comprendre, dans la mesure où le projet d'enfant est, aujourd'hui encore, source de discrimination dans le monde de l'entreprise. Mais nous croyons qu'il est indispensable de leur laisser le choix de prendre

les fausses couches peuvent être vécues comme traumatisantes, ou en tout cas avoir des conséquences psychologiques lourdes. Dès lors, proposer un congé spécifique pour fausse couche, c'est être à la hauteur de la douleur physique et psychologique liée à l'échec à l'échec du projet d'enfant ; créer ce congé, c'est créer un droit automatique qui n'a pas à être négocié, qui peut être choisi ou écarté, mais qui représente une liberté et une protection pour les femmes.

Or révéler son interruption spontanée de grossesse à son employeur pourrait, bien malheureusement, exposer les personnes qui y sont confrontées à des discriminations supplémentaires, pour raisons familiales, en dévoilant un désir réel ou supposé de parentalité. La commission a exprimé sa préoccupation pour l'égalité professionnelle, qui passe ici par la garantie de la discrétion professionnelle, comme l'ont révélé les auditions que nous avons conduites. En ce sens, il nous apparaît précipité de généraliser ce congé dès aujourd'hui.

? Bien sûr, vivre une interruption spontanée de grossesse est une épreuve pour la femme et pour le couple, une épreuve qui peut susciter un temps d'arrêt de travail. Il n'est pas opportun de figer

est arrêtée. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important en matière d'égalité professionnelle : la femme doit rester libre d'informer son employeur d'une grossesse en cours ou d'un projet de grossesse, En complément de ce nouveau dispositif légal, les partenaires sociaux peuvent, par accord collectif, marquer leur volonté de contribuer au développement d'un environnement de travail permettant une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie entre vie professionnelle et vie personnelle. Ils ont un rôle à jouer en tant qu'acteurs clés de cette conciliation. On constate aussi que les entreprises investissent davantage les thèmes de la parentalité et des aidants. Il faut saluer ces initiatives et faire confiance aux partenaires sociaux. Pour l'ensemble de ces raisons, je suis défavorable à ces amendements.

Le scrutin est clos.

que des discriminations associées au désir réel ou supposé de parentalité qu'elle peut révéler à l'employeur, une telle protection apparaît justifiée. L'adoption de cet amendement permettra également de rapprocher le droit applicable aux fausses couches tardives de celui qui régit de nombreuses situations ayant trait à la grossesse ou à la perte d'un foetus pour lesquelles la loi prévoit déjà des protections contre le licenciement : grossesse, naissance récente, congé maternité, ou encore perte de grossesse après la 22 semaine. Il revient Il revient donc bien ici à la loi de compléter les protections existantes afin de limiter les effets de seuil : aujourd'hui, une grossesse arrêtée à 22 semaines d'aménorrhée moins un jour

un avis favorable de la commission.

L'association dénonce le manque d'information à l'école et de vulgarisation scientifique, responsable de la culpabilisation des femmes qui subissent une perte de grossesse précoce, autant que du passage sous silence de cet événement- et, nous venons de le voir, cela ne va pas s'améliorer.

de la commission ? Je partage pleinement le constat qui sous-tend cet amendement : l'information et la sensibilisation autour des interruptions spontanées de grossesse sont largement insuffisantes.

En effet, les séances d'éducation à la sexualité, dont le programme- déjà particulièrement chargé -inclut la sexualité, les violences sexistes et sexuelles et les mutilations sexuelles, n'ont pas été pensées pour englober, au surplus, les divers aspects de la grossesse. de former les élèves, dans une approche moins académique, à la découverte de la vie sexuelle, que tous ne peuvent pas sereinement aborder à la maison. L'interruption spontanée de grossesse gagnerait plutôt à faire l'objet d'une formation académique, intégrée dans les programmes de sciences de la vie et de la terre au collège, puis au lycée. Une telle formation, plus rigoureuse scientifiquement, semble mieux à même de répondre aux idées préconçues inexactes qu'évoque le collectif « Fausse couche, vrai vécu » dans sa tribune. Les programmes scolaires relevant du domaine réglementaire, il appartiendra au ministre de l'éducation nationale de saisir le Conseil supérieur des programmes pour étudier l'opportunité de renforcer la place qui y est consacrée aux interruptions spontanées de grossesse. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Madame la ministre,

tous les thèmes à la fois de la sexualité et de la reproduction.

le ou la » partenaire. C'est d'ailleurs en ces termes que le ministre de la santé s'est exprimé devant les députés le 8 mars dernier, déclarant : « Grâce Grâce à cette future loi, les sages-femmes seront désormais habilitées, dans tout type de situation liée à la grossesse, à adresser leurs patientes à ce dispositif d'accompagnement psychologique. S'il s'agit d'une fausse couche, le ou la partenaire de la patiente pourra également en bénéficier, toujours par l'intermédiaire de la sage-femme. » Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec le ministre de la santé- c'est à noter. C'est un scoop ! Aussi, je pense que Martin Lévrier ne peut que me suivre

Poncet Monge Il s'agit d'un amendement de Mélanie Vogel. Faciliter l'accompagnement psychologique après une fausse couche constitue une avancée que nous saluons.

dans un désert médical, où un accès à un psychologue est difficile. C'est pourquoi nous demandons de rembourser l'accompagnement psychologique dans un désert médical, même si la première séance s'est tenue en

de la commission ? Le code de la santé publique permet déjà la réalisation des séances par vidéotransmission, à l'exception de la première séance, qui est consacrée à un entretien d'évaluation. Il me semble que cette mesure permet un équilibre pertinent entre accès aux soins et qualité de l'accompagnement psychologique. De plus, il ne paraît pas souhaitable de prévoir des règles différentes en la matière, selon que le trouble psychologique est consécutif à une interruption spontanée de grossesse ou non. En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

présenter l'amendement n° 2 rectifié. Le dispositif MonParcoursPsy a été lancé le 5 avril 2022 pour lutter contre les effets psychiques de la crise sanitaire. Un an plus tard, nous ne pouvons que constater que le bilan est plus que mitigé : seulement 90 000 patients ont bénéficié du dispositif et moins de 10 % des ont adhéré au système, 93 % environ le refusant, pour de multiples raisons. L'objectif de cette proposition de loi est bien de garantir aux femmes confrontées à une interruption spontanée de grossesse un suivi médical, mais surtout un suivi psychologique, qui repose en grande partie sur l'efficience de MonParcoursPsy.

Nous pourrions penser que nous avons tous pris conscience de l'importance de lever le non-dit et de consacrer des mesures fortes pour accompagner les couples confrontés à une interruption de grossesse. Pourtant, nous empêchons souvent des avancées qui amélioreraient l'accompagnement des femmes et de leur partenaire.

déjà aux professionnels de santé. Or force est de constater que, si cette obligation existe, elle n'est pas respectée par certains professionnels de santé. Dès lors, le rapporteur doit soit proposer de renforcer les sanctions en cas de non-respect de leur obligation,

En tout état de cause, nous proposons, par cet amendement, d'améliorer la reconnaissance de l'interruption spontanée de grossesse et de garantir une prise en charge médicale adéquate des femmes qui en sont victimes. Il s'agit donc réellement d'un amendement d'amélioration, qui prend en considération le travail de l'Assemblée nationale.

que, s'il y a une « fausse couche », la grossesse a bien existé et doit être prise en charge par la sécurité sociale. C'est aussi moins protéger la femme enceinte puisque, avant six mois de grossesse, de grossesse, tout arrêt, hors fausse couche, on l'a vu aujourd'hui, devenant un simple arrêt maladie, occasionne des jours de perte de salaire, alors que le droit du travail reconnaît que, dès le quatrième mois de grossesse, la femme doit bénéficier d'une protection, à savoir la réduction du temps de travail.

toutefois une grossesse. C'est pourquoi cet amendement a pour objet la remise d'un rapport sur la possibilité d'étendre l'assurance maternité. Votre

un avis défavorable sur cet amendement. La couverture maladie des risques associés à la maternité intervient dès le début de la grossesse. Elle permet de prendre en charge les examens médicaux obligatoires dans le cadre du suivi de grossesse, notamment en cas de grossesse pathologique ou de pathologie foetale. Dans la pratique, il serait impossible d'étendre cette prise en charge par la maternité avant même la déclaration de grossesse, qui doit intervenir avant la fin du troisième mois. C'est C'est dans le cadre du premier examen prénatal que le professionnel de santé- médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme -procède à la déclaration de grossesse et la signale à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. À partir de cette information, la caisse déclenche la prise en charge au titre de la maternité. Il semble nécessaire de maintenir le partage entre prise en charge du risque maladie et prise en charge du risque maternité. Je mets aux voix l'amendement

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert.

Le scrutin est clos.

à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes ; Conclusions de